réserves d'usage. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Georges Dessaigne, qui fut sénateur de la Mayenne de 1986 à 1988 puis de 1995 à 1997, et Jacques Bimbenet, qui fut sénateur de Loir-et-Cher de 1986 à 2001. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la délibération de la commission mixte paritaire a été conclusive. Nous sommes donc arrivés à un accord sur un projet de texte partagé entre députés et sénateurs.

Mme la ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, après que l'Assemblée nationale a adopté, le 14 mai dernier, les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, il appartient aujourd'hui à la Haute Assemblée de se prononcer sur le résultat des travaux de cette commission, afin de mettre un terme à ce processus parlementaire entamé il y a maintenant plus de six mois. Je veux bien entendu, au nom du Gouvernement, me féliciter de l'accord auquel sont parvenus les députés et les sénateurs lors de la réunion de la commission mixte paritaire le 18 avril. Qu'il me soit permis, à cet égard, de remercier et de féliciter votre rapporteur, M. Alain Richard, pour la qualité de son travail et son sens de l'écoute et du compromis, qui ont été précieux pour le bon aboutissement, si vous en décidez ainsi dans quelques instants, de ce texte. Je veux Je veux également remercier l'ensemble des sénateurs qui se sont mobilisés lors de l'examen du projet de loi et qui, par-delà la diversité de leurs sensibilités politiques, se sont réunis pour apporter une majorité à l'approbation de cette réforme électorale importante. J'ai évoqué un processus législatif déjà long de six mois puisque, en amont même de l'adoption du texte en conseil des ministres,

ces discussions, le Gouvernement a estimé qu'une solution s'imposait : le rétablissement d'une circonscription nationale. Au demeurant, la plupart des formations politiques consultées préalablement au passage du texte en conseil des ministres en ont convenu. D'ailleurs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, vous en avez aussi convenu, puisque vous avez, à une large majorité, adopté le rétablissement de la circonscription unique. Ce système nous rapproche de nos partenaires européens,

Le Gouvernement est convaincu que cette option était la seule à même de garantir un intérêt accru des électeurs pour ce scrutin, en élevant au niveau national le débat autour des grands enjeux européens. Au-delà de cette réforme inscrite dans le projet de loi et des conséquences législatives qu'il convenait d'en tirer dans la loi du 7 juillet 1977, nous étions tenus de faire évoluer les dispositions relatives à la répartition du temps d'antenne

dans sa décision du 31 mai 2017. Initialement, le Gouvernement avait proposé un dispositif reposant sur un triple mode de répartition : un temps forfaitaire ; une durée de deux heures répartie en fonction du nombre de députés et de sénateurs ; enfin, une dernière fraction à vocation corrective. Alors que le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait que le résultat des dernières élections européennes serait pris en compte dans la troisième fraction corrective, vous avez décidé, sur proposition de votre rapporteur, que le temps réparti entre les listes au titre de la deuxième fraction prendrait en compte, au-delà du nombre de députés et de sénateurs déclarant soutenir ces listes, le nombre de députés européens.

Sur ce même article, le Gouvernement se réjouit que la commission mixte paritaire ait trouvé un compromis quant aux modalités de fonctionnement de cette fraction à vocation corrective : à la marge de manoeuvre donnée par le Sénat au CSA de choisir une durée à répartir comprise entre une heure et une heure trente- dispositif dont le Gouvernement craignait qu'il encoure le risque d'être censuré pour incompétence négative du législateur -, il a été préféré un dispositif portant la troisième fraction à une heure trente, ce qui apparaît plus satisfaisant sur le plan juridique et opérationnel. Enfin, le dernier point sur lequel les deux assemblées avaient une différence d'appréciation était l'article 7, en ce qu'il faisait référence à l'élection de députés européens sur des listes transnationales dans le cadre d'une circonscription européenne unique, référence qui avait été supprimée lors de l'examen du texte Tout en prenant acte du vote négatif du Parlement européen en février dernier, le Gouvernement reste très engagé dans la poursuite des négociations européennes et continuera à défendre cette idée, car elle est, de notre point de vue, l'un des axes majeurs de renforcement de la démocratie européenne. Cette proposition, soutenue par bon nombre de nos partenaires, continue de faire l'objet de négociations dans la perspective des futurs scrutins européens. C'est pourquoi le Gouvernement exprime sa satisfaction que la commission mixte paritaire

collègues, les membres du groupe du RDSE voteront, sans réserve, pour l'adoption de ce projet de loi, qui permet un retour à la circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Comme nous le faisons valoir depuis 2010, rien ne permet de dire que le découpage en huit circonscriptions a atteint les objectifs fixés par la loi de 2003. Constatant que le lien entre l'électeur et l'élu se trouve excessivement distendu, celle-ci visait à faire sortir les élus de « l'anonymat des listes nationales

parfois totalement opposés. C'est la preuve qu'on ne peut se rattacher à des sentiments pour évaluer ce lien de proximité. Le seul fait objectivement mesurable est l'abstention. Or, comme vous le savez tous, l'abstention aux élections européennes n'a cessé de croître. Je ne reviendrai pas non plus en détail sur les conditions d'adoption du découpage actuel et le recours à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par le Gouvernement de l'époque, qui soulignait l'importance politique de la question. En effet, bien que le législateur s'en soit expressément défendu en 2003, le découpage en huit circonscriptions a contribué à affaiblir les effets du scrutin à la proportionnelle. Au moment de son adoption, ce choix était justifié par le rôle marginal du Parlement européen, qui servait de faible décorum démocratique. Comme le rappelait l'exposé des motifs de la de 2003, « cette consultation, eu égard aux compétences du Parlement européen, n'a pas pour objet de dégager une majorité de Gouvernement. Dans ces conditions, le législateur a estimé souhaitable de faire en sorte que toutes les sensibilités politiques puissent être représentées au Parlement de Strasbourg ». Il est clair que le traité de Lisbonne, en modifiant les équilibres institutionnels européens, a rendu ce raisonnement caduc, sans effacer l'impératif de représentativité au sein de l'Union européenne. Les débats autour de la désignation du président de la Commission européenne et de la règle des impliquent au contraire de renforcer la légitimité de nos représentants au Parlement européen. Nous restons convaincus que le rétablissement de la circonscription unique remédie à la marginalisation électorale de ces représentants. Il pourrait également renforcer leur mandat, en leur donnant une légitimité plus forte, proportionnelle à leur base électorale, et consolider ainsi leur poids dans les négociations quotidiennes avec leurs collègues européens. Pour autant, nous n'avons pas la naïveté de croire que ce texte permettra à lui seul de restaurer un lien de qualité entre les Français et leurs élus au Parlement européen. Nos principaux amendements tendaient d'ailleurs à souligner l'important travail de pédagogie à conduire sur le rôle croissant du Parlement européen au sein des institutions européennes. Ces propositions s'inscrivaient totalement dans l'esprit du discours de la Sorbonne du Président de la République, dans lequel il déclarait : « Organisons un débat ouvert, libre, transparent, européen, pour construire ce projet qui peut donner enfin un contenu et un enjeu à nos élections européennes de 2019. Une plus grande médiatisation des sujets européens reste absolument nécessaire, en parallèle des consultations européennes organisées par le Gouvernement. Comme je le disais, nous adopterons ce texte sans réserve, mais avec quelques regrets Malgré cela, nous nous félicitons des arbitrages retenus par la commission mixte paritaire sur la rédaction des articles 2 et 2 , qui permettront d'apporter un peu plus de réalisme dans des règles de calcul de temps de parole relativement complexes. En particulier, la solution proposée par notre rapporteur d'allonger le temps de parole réparti par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une heure à une heure trente présente le double avantage d'augmenter la durée totale des débats consacrés à l'Union européenne et de faciliter les péréquations. La prise en compte de la représentativité des listes nationales en fonction du soutien apporté par des députés et sénateurs, mais également par des membres du Parlement européen, est plus pertinente au regard de l'objet du texte. Il aurait été paradoxal que le temps d'antenne accordé aux candidats aux élections européennes reste principalement déterminé par la représentativité de leur mouvement politique au niveau national. Il ne faut pas minimiser les défis qui attendent les futurs membres du Parlement européen. Le changement de découpage électoral présente un enjeu important, qui a été très débattu au moment de l'examen de l'article 1, à propos de la représentation des territoires d'outre-mer. Le droit de l'Union européenne étant plus attaché à la différenciation territoriale que ne l'est le droit français, nos prochains représentants au Parlement européen devront être particulièrement vigilants Enfin, et c'était le sens de notre soutien au développement de listes transnationales, il reviendra à nos représentants de faire émerger de véritables formations politiques européennes et de promouvoir le parlementarisme au sein de l'Union pour y apporter toute la représentativité que nos concitoyens attendent. La parole

aux élections européennes constitue un réel problème et est préjudiciable à la démocratie. Il est nécessaire que les citoyens adhèrent à l'idée européenne, et je suis intimement convaincue qu'on ne fait pas le bonheur des peuples malgré eux.

et ne résoudra finalement ni le problème de l'abstention ni la crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les citoyens et l'Europe. C'est pourquoi le groupe Les Républicains s'opposera au texte tel qu'il est proposé aujourd'hui.

résultat ! La majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat se sont accordées dès la fin de la première lecture sur une rédaction de ce projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, mais aussi aux élections législatives- il faut le rappeler ! nous estimons positif le retour à la circonscription unique pour l'organisation du scrutin, nous regrettons plusieurs dispositions que nous jugeons particulièrement négatives. critiqué fortement la régionalisation du scrutin européen, affichée comme un moyen de répondre à la baisse de la participation, mais qui répondait, selon nous, à une volonté de régionalisation de l'Europe elle-même, ainsi qu'à l'objectif de bipolarisation de la vie politique, car les deux principales formations d'alors espéraient être favorisées, tout en écartant les listes plus minoritaires. Même si nous n'avons pas d'éléments précis, accordons-nous sur l'idée que les circonscriptions régionales ont été un échec, puisque l'abstention s'est fortement accrue depuis 2004, comme je le démontrais lors de mon intervention en première lecture le 10 avril dernier. Nous approuvons donc ce retour à la circonscription unique, sans pour autant être dupes du choix politicien du Président de la République, qui souhaite user d'une liste unique pour faire prévaloir sa puissance de feu médiatique qui palliera sans doute les défaillances du mouvement La République En Marche sur le terrain. Deux points du texte issu de la commission mixte paritaire suscitent toujours notre opposition. Premièrement, nous regrettons fortement le maintien d'un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour participer à la répartition des sièges. Ce seuil, que seuls neuf pays européens ont adopté, porte un coup au pluralisme. Ainsi, une liste recueillant plusieurs centaines de milliers de voix, voire largement plus de un million en cas de participation plus élevée, ne pourra pas être représentée au Parlement européen. C'est un véritable Aucun argument sérieux n'a été apporté au cours de la discussion pour justifier un tel ostracisme à l'égard de plusieurs courants de pensée dans notre pays. Au minimum, pourquoi ne pas avoir harmonisé ce seuil de 5 %

ce point est bien lié au précédent, nous sommes opposés à la modification des règles de la campagne audiovisuelle, qui, en substituant au principe d'égalité celui d'équité, favorisera, malgré les- faibles -dispositifs de pondération, les partis dominants, à commencer par celui du Président de la République. le Gouvernement a profité de ce texte, un amendement déposé en pleine séance à l'Assemblée nationale, pour modifier dans le même sens les règles de la campagne audiovisuelle pour les élections législatives. Il me semble que la précipitation n'est pas un bon choix pour un élément essentiel du débat politique. Enfin, un troisième point

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, simplicité et gravité sont les deux mots qui me viennent à l'esprit en prenant la parole devant vous ; simplicité sur la forme, gravité sur le fond.

il devenait cohérent qu'un accord soit trouvé entre les deux chambres. La commission mixte paritaire du 18 avril a été positive, ce dont je me réjouis avec mes collègues du groupe Union même si la dimension ultramarine de notre groupe ne se satisfait pas de la circonscription électorale unique, comme vous en fera part notre excellent collègue Gérard Poadja. Si le sujet électoral est simple, la question de fond pousse à plus de gravité.

par les Européens. Ces sanctions, décidées par un seul pays, s'appliqueraient aux entreprises d'autres pays, notamment le nôtre. C'est dire, chers collègues, que la poursuite de l'approfondissement de la construction européenne est au coeur de notre combat politique, de ce que nous souhaitons pour notre pays.

et les tensions de toutes sortes pour conforter leur autorité politique. Trop de pays, y compris en Europe, au motif d'efficacité, de souveraineté populaire, s'écartent des valeurs démocratiques, de la liberté de la presse ou de l'indépendance de la justice. L'unilatéralisme fait rage, là où notre pays a toujours pensé que les États étaient interdépendants et que les bons accords étaient multilatéraux et non de vainqueurs à vaincus.

L'accessoire, c'est le mode électoral que nous allons utiliser en 2019. L'essentiel, c'est la manière dont notre pays sera capable de se rassembler pour exprimer de la manière la plus unitaire possible notre parole en Europe,

Les listes nationales le permettront mieux. Les listes transnationales le permettraient plus encore. Les listes transnationales- puisque tel est le sujet de l'article 7 -permettraient aussi aux partis, aux

en dépit des bourrasques, dont le Brexit, la crise migratoire et les élections italiennes sont les plus récentes. Elle parvient- plus souvent qu'on ne le dit et n'en déplaise à ses détracteurs -à décider j'en veux pour preuve, par exemple, le déclenchement de la loi de « blocage » par la Commission vendredi pour protéger nos entreprises opérant en Iran des sanctions américaines. Dans un an, en mai 2019, l'Union européenne connaîtra un moment important : nous devrons choisir entre une Europe qui décide ou une Europe qui subit. Pour la neuvième fois depuis 1979, 500 millions de citoyens européens seront appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants au Parlement, l'instance qui constitue non seulement l'organe législatif de l'Union européenne, mais également- et surtout -le lieu central de l'expression démocratique européenne. Or, malgré cette élection au suffrage universel direct, le niveau de participation électorale aux scrutins européens a chuté de 46,8 % en 1999 à 42,4 % en 2014. en huit circonscriptions issu de la réforme du 11 avril 2003 visait à susciter l'intérêt de l'électorat français pour les élections européennes et à resserrer les liens démocratiques entre les citoyens et leurs élus. Il faut bien reconnaître qu'il a échoué. Ce découpage ne correspond à aucune réalité concrète : il manque de cohérence historique, culturelle, économique, sociale et administrative. Il nous éloigne du modèle majoritaire de circonscription unique retenu par vingt-deux des vingt-sept États membres. Les circonscriptions interrégionales doivent demeurer l'exception, parfois justifiées par l'existence d'un État fédéral comme en Belgique ou en Italie. Avec ce projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, il s'agit, pour l'essentiel, de rétablir le principe de la circonscription unique. La circonscription nationale apparaît la plus conforme à la nature de l'élection européenne et surtout la plus à même de faire de nos représentants les mandataires de la nation française tout entière. Je me réjouis donc que le territoire de la République soit considéré comme une circonscription unique. Cependant, une attention particulière devra être portée, lors de la composition des listes, à une représentation équilibrée de tout le territoire, notamment du monde rural et des outre-mer. Dans la réalité de la configuration actuelle, seuls les principaux bassins de vie bénéficiaient de la présence d'un député européen, et les territoires ruraux étaient, de fait, souvent mis de côté. Je souhaite également saluer les dispositions relatives à l'organisation de la campagne des élections européennes à la radio et à la télévision, ainsi que celles qui sont relatives à la transparence des dépenses électorales engagées par les partis et groupements politiques en soutien d'une liste de candidats aux élections européennes. Ces mesures participent à la modernisation de la vie politique. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire ait abouti à un accord sur un texte qui procède d'une ambition forte, celle de replacer l'Europe au coeur de la vie démocratique de notre pays. J'espère que ce texte contribuera à rendre le débat européen plus présent et plus visible aux yeux de nos concitoyens en permettant non seulement de mettre les grands dossiers de la politique européenne au premier plan des discussions, mais également de forcer chacune des forces politiques françaises à prendre clairement position. Madame la ministre, mes chers collègues, ma génération s'est engagée pour l'Europe. Ma génération croit à l'Europe, parce qu'elle a compris les effets de son absence : la guerre ou la peur de la guerre, la misère et la haine. Toutes les générations avant la mienne, avant la nôtre, ont eu à l'esprit une guerre qu'elles devaient subir ou à laquelle elles devaient participer. La nôtre est la première qui n'a pas connu cette fatalité, et nous devons oeuvrer pour que cela perdure. Nous en avons le devoir envers notre jeunesse et les générations futures. fondée sur la volonté de vivre et de progresser en commun, porteuse d'espérance et tournée vers l'avenir, l'Europe est une promesse de paix, de prospérité et de liberté. Elle est un désir de fraternité. raison pour laquelle la diminution de la participation électorale à laquelle les gouvernements successifs se sont habitués ne doit pas nous laisser indifférents. Bien au contraire, adopter toutes les mesures indispensables au renforcement de la légitimité et de la représentativité du Parlement européen apparaît plus que jamais nécessaire.

les territoires d'outre-mer, lesquels risquent de voir leur représentation insuffisamment prise en compte. Ce sera la responsabilité des auteurs des listes présentées de prendre leurs décisions en ce domaine.

Madame la présidente, madame le ministre, chers collègues, dans ce texte, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est le retour

Les découpages par pseudo-régions européennes n'avaient absolument aucun sens. Pour moi qui suis un ancien, je peux dire que, l'objet de ces découpages, c'était d'affaiblir l'effet de la proportionnelle. En gros, il s'agissait à l'époque d'une opération politique menée par des partis qui n'avaient pas de bonne tête de liste et qui voulaient avoir des sous-listes régionales, ce qui permettait de magouiller un petit peu et d'éviter une expression forte

parce que c'est la France qui doit s'exprimer, il est tout aussi scandaleux de vouloir faire des listes supranationales qui amputeraient- et c'est l'article 7 que je vise ici ! -la souveraineté nationale et la force de notre pays au sein de l'Union européenne. Avec mes deux collègues

qui fait allusion aux listes supranationales. D'ailleurs, en commission, j'avais moi-même déposé un amendement qui anticipait en proposant de supprimer la phrase correspondante,

Je ne comprends pas que le Gouvernement, qui se plaint tout le temps de ce que le Parlement ne cesse d'ajouter des textes qui ne servent à rien et qui ne sont pas législatifs, donne le mauvais exemple. Je le dis très clairement le Gouvernement donne un mauvais exemple ! C'est la raison pour laquelle, bien que je sois pour le texte,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer ici le travail très constructif de la commission mixte paritaire qui s'est tenue la semaine passée. Il a permis d'aboutir à un à un accord sur la base d'un texte très proche de celui que nous avions adopté lors de sa première lecture au Sénat, le 10 avril dernier. Ce type de situation n'est pas si fréquent. Nous aurions donc tort de ne pas nous en réjouir, car cela souligne bien l'assez large consensus au sein de la représentation nationale quant à un retour à la circonscription unique pour la désignation de nos représentants au Parlement européen. Tout cela est, somme toute, assez logique au regard du fait électoral. Le découpage du territoire national en huit eurocirconscriptions, qui a présidé à la tenue de ce scrutin en France lors de ses trois dernières éditions, n'a en effet pas tenu ses promesses initiales, au premier rang desquelles celle de provoquer une participation accrue du corps à l'occasion d'une élection dont les enjeux n'ont pourtant jamais été aussi prégnants. Ce retour à la circonscription unique provoquera-t-il un sursaut de participation chez nos concitoyens

Très sincèrement, nous le croyons ! D'abord, parce qu'il offrira plus de lisibilité aux enjeux européens et plus de visibilité et de clarté aux propositions politiques des différentes listes qui seront en lice. De fait, la répartition des sièges sera plus équitable au regard des suffrages obtenus par chacun des compétiteurs. Rappelons qu'il fallait jusqu'à présent recueillir au moins 15 % des suffrages exprimés dans la région Massif central-Centre pour espérer obtenir un siège quand il suffisait de franchir le seuil des 5 % en région Ile-de-France pour en gagner un ! Il y aura donc plus d'équité entre les électeurs de nos différents territoires, et c'est une chose importante, mais également plus de lisibilité. En effet, nous éviterons la démultiplication extrême des listes en compétition plus d'une quarantaine en 2014 en raison du nombre élevé- plus de la moitié -de celles qui ne concourraient que dans une ou deux eurocirconscriptions seulement, lesquelles, comme par hasard, étaient les plus dotées en sièges à pourvoir. Ce retour à la circonscription unique ainsi que le mode de répartition plus équitable du temps de parole proposé par ce texte suffiront-ils à générer une plus forte implication des électeurs à l'égard des élections européennes ? Une chose est certaine, c'est qu'ils y contribueront. Nous ne sommes cependant pas naïfs au point de penser que les choix normatifs entourant les modalités de scrutin suffisent à entraîner l'enthousiasme participatif de citoyens souvent blasés des postures politiciennes et des promesses non tenues. Le reste du chemin à parcourir pour faire venir ou revenir les électeurs vers les urnes relève aussi, et peut-être avant tout, des choix politiques qui seront opérés par les formations et les listes qui candidateront. Va-t-on, contrairement à ce qui s'est souvent fait par le passé, mettre enfin la question européenne réellement au coeur de la campagne, plutôt que de transformer systématiquement cette élection en un petit tour de chauffe d'une élection présidentielle présidentielle toujours à venir ? Le scrutin de liste a ses qualités et ses défauts. Il a aussi, pour certains, le défaut de ses qualités. Il renvoie clairement aux formations politiques la responsabilité du choix et de l'ordonnancement des candidats qui concourront en leur nom. Ce sont à à elles que revient en effet cette responsabilité, celle de présenter des candidats compétents, issus des différents territoires et qui s'investiront pleinement dans leurs fonctions d'eurodéputés. Il est de bon ton, en France, de présenter les élections européennes comme un scrutin permettant de recaser un tel ou un tel pour service rendu ou d'exfiltrer élégamment telle ou telle personnalité devenue encombrante dans l'arène politique nationale. Ça peut arriver ! Vous savez de quoi la faute, sinon auxdites formations politiques ? On vante aussi souvent, en France, la très forte implication et l'influence exercée par certaines délégations nationales au sein du Parlement européen, notamment la délégation allemande. Pourtant, elles sont presque toutes élues dans le cadre d'une circonscription unique. On le voit bien, c'est la conjonction de normes justes et efficientes et de bonnes pratiques politiques, jusqu'au sein de nos propres formations, qui font la vitalité de notre démocratie et de sa représentation. ce n'est pas de déplorer, au soir de chaque élection, un nouveau recul de la participation, mais bien de se livrer régulièrement à une évaluation rigoureuse des choix, tant législatifs que politiques, auxquels nous avons procédé pour mobiliser le plus grand nombre. C'est précisément ce type d'évaluation des trois derniers scrutins européens en France qui nous conduit à soutenir le retour à la circonscription unique et à vouloir créer les conditions d'un véritable débat national sur l'avenir de l'Europe. Le bon sens tout court- et pas seulement le bon sens politique -devrait nous amener de la même manière à procéder, à l'issue des prochaines élections européennes, l'année prochaine, à une nouvelle évaluation des effets des mesures proposées dans ce texte. C'est parce que nous avons la conviction profonde que celles-ci devraient nous permettre d'enrayer l'insupportable désertion des urnes, à un moment où l'Union européenne est à refonder pour continuer d'exister,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous discutons une nouvelle fois, dans cet hémicycle, du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, texte qui nuit à la représentation de la population française, notamment dans ses dimensions ultramarines. En effet, dans le cadre du dispositif électoral aujourd'hui en vigueur, la circonscription outre-mer est constituée de trois sections : Atlantique, océan Indien et Pacifique. Depuis 2009, pour la première fois dans l'histoire de la représentation française au Parlement européen, les outre-mer de chaque océan avaient donc la garantie de disposer d'un représentant à Bruxelles. Le choix qu'a fait le Gouvernement d'une circonscription électorale unique conduit inéluctablement la diversité ultramarine à ne plus pouvoir s'exprimer au Parlement européen, car la représentation des outre-mer est désormais soumise au bon vouloir des partis politiques. Or, lorsque les partis politiques témoignent de leur attachement aux outre-mer, l'arithmétique électorale étouffe les collectivités les moins peuplées, au premier rang desquelles celles du Pacifique. européennes de 1999 en ont constitué une illustration caricaturale, avec l'élection au Parlement de trois Ultramarins qui, bien qu'issus de trois listes politiques différentes, étaient tous les les trois de La Réunion. J'en profite pour saluer mes collègues Réunionnais, département ultramarin comptant le plus d'électeurs. Je suis d'autant plus atterré par le mode de scrutin retenu que l'étude d'impact demandée pour ce projet de loi affirme, de manière mensongère, que « le le maintien d'une circonscription ultramarine serait susceptible d'engendrer pour les populations outre-mer le sentiment de bénéficier d'un traitement politique différencié auquel elles n'aspirent pas nécessairement À la lecture de ces lignes et constatant les prises de position de mes collègues Ultramarins sur ce texte, j'en viens à me demander d'où sort cette affirmation. Il faut un référendum ! Nous voulons justement pouvoir faire valoir notre diversité notre diversité et défendre nos spécificités à l'égard de l'Union européenne. Madame la ministre, qui mieux qu'un habitant des outre-mer pour défendre les intérêts de sa région ? région ? Enfin, ce texte ne s'inscrit pas dans la perspective pour le Pacifique tracée par le Président de la République lors de son discours au théâtre de l'Île, à Nouméa, le 5 mai dernier, au cours duquel il a exposé « la stratégie indopacifique » que la France et l'Union européenne doivent développer à travers l'axe Paris-New Delhi-Canberra-Nouméa-Papeete. Le chef de l'État a notamment insisté sur un fait politique majeur après le Brexit, la France « devient le dernier pays européen du Pacifique » grâce à ses trois territoires : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Madame la ministre, après l'adoption de ce projet de loi, le Pacifique deviendra le grand oublié des outre-mer français au Parlement européen, au moment même où l'État est engagé dans la défense des intérêts des PTOM, leurs statuts devant être renégociés dans la perspective de la fin des accords de Cotonou en 2020. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est avec une grande déception que je voterai contre ce projet de loi, comme l'ont fait à l'Assemblée nationale mes collègues députés du Pacifique.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

si ce dernier a été passé illégalement. Devant ce risque, les responsables des marchés rechigneraient à utiliser les possibilités de procédures simplifiées, en particulier les marchés de gré à gré sans mise en concurrence. Cette difficulté, il nous faut la résoudre collectivement.

et de montrer aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie dans nos armées que nous faisons tout ce qui est possible pour les doter des meilleurs équipements et des meilleurs matériels, que ce soit pour affronter l'ennemi ou pour assurer leur propre protection contre celui-ci.

Au-delà du débat sur les surtranspositions, sur lesquelles vous souhaitez revenir, madame la ministre, mais auxquelles vous ne voulez pas que le Sénat touche, se pose plus généralement la question des conditions dans lesquelles nos armées s'équipent. Les sujets sont multiples et difficiles, et nous en avons des exemples divers et variés. Il y a, bien sûr, la confidentialité des informations- et notre ajout en commission y a trait. Il y a la lenteur et la lourdeur des procédures, qui sont souvent à la fois inadaptées aux besoins nouveaux identifiés en opération et porteuses du risque d'obsolescence des matériels livrés, à un moment où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts et où il faut acheter vite pour être efficace. Il y a l'absurdité- il faut bien nommer les choses -d'une pratique qui consiste à devoir requalifier des matériels qui sont en service depuis des années dans les armées de pays amis et proches,

que sénatrices et sénateurs, nous sommes engagés dans la vie publique, au service de notre pays, mais nous ne risquons pas notre vie et n'avons nul besoin de tels matériels. Comment expliquer à nos soldats qu'il faille attendre parfois des années pour un équipement permettant de faire face aux adversaires qu'ils rencontrent sur le terrain ? Je rappelle aux esprits adeptes des subtilités du droit que, pour l'instant, les groupes terroristes n'ont pas choisi d'appliquer le code des marchés publics. Si notre droit ne permet pas d'acheter dans des conditions raisonnables les matériels nécessaires- je ne parle pas des programmes à effet majeur -, eh bien, changeons-le ! Dans cette perspective, il va de soi que nous vivons mal l'amendement du Gouvernement visant à supprimer le dispositif voté par la commission la semaine dernière. Je soupçonne la DGA de faire un peu de lobbying

seuls l'État et ses établissements publics peuvent conclure des marchés de défense et de sécurité. La seconde condition est matérielle : les marchés de défense et de sécurité sont ceux

observations sur une subtilité qui ne nous paraissait pas aussi claire. Pour autant, nous maintenons cet amendement. Nous en reparlerons lors de la commission mixte paritaire.

un certain nombre de cas de dispenses des règles de publicité et de mise en concurrence qui sont spécifiques au marché de défense et de sécurité. Dit ainsi, cela paraît très abstrait. En réalité, la disposition introduite par la commission correspond à une préoccupation, que je partage pleinement, qui consiste à essayer d'exploiter au mieux toutes les marges de manoeuvre offertes par le droit européen en vue de faciliter les acquisitions les plus sensibles du ministère des armées. Si nous partageons la philosophie Si nous partageons la philosophie qui motive cette disposition,

intègre dans l'ordonnance des illustrations de ce que pourrait recouvrir chacun des cas d'exclusion. Cela présente de sérieux risques, les les illustrations qui ne sont pas citées pouvant être considérées comme ne pouvant donner lieu à exclusion du champ de l'article.

élargissant le champ d'application des différentes exclusions à la procédure de mise en concurrence prévue par la directive. Au-delà de ces aspects strictement juridique et rédactionnel, je précise

de rendre les acquisitions d'un certain nombre de services de forces, en particulier ceux qui ont besoin d'expérimenter du matériel sur des petites séries. Nous pouvons y parvenir dans le cadre d'une instruction sur laquelle nos services travaillent actuellement et qui permettrait aux services acheteurs d'utiliser au mieux toutes ces souplesses, ce que, en effet, ils ne font pas aujourd'hui.

d'information de notre assemblée signé par Gérard Larcher, Jacques Gautier et Daniel Reiner pointait déjà le fait que nombre de procédures d'acquisition ne convenaient absolument pas dans un certain nombre de cas, notamment pour les forces spéciales ? Il faut aborder

Contrairement à ce que vous avez affirmé, il ne s'agit pas simplement de transposer un considérant- ce serait en effet juridiquement assez étrange. Il s'agit d'user des facultés que nous donne la directive européenne, dont je dois rappeler qu'elle a été négociée sous présidence française et que la France était alors très

Il est vrai qu'actuellement la loi promeut une transparence totale en matière de passation de marchés publics. C'est logique : il s'agit de l'argent du contribuable et d'une question d'intérêt général ; mais il est tout aussi vrai que la défense n'est pas n'importe quel secteur et que le secret relève parfois de la sécurité nationale.

En effet, il existe de véritables enjeux en matière de marchés publics de défense : montants concernés, présence d'intermédiaires et des commissions afférentes, domaines sensibles. Ces sujets concernent l'ensemble de la communauté nationale. C'est dans cette recherche d'équilibre que s'inscrit cet amendement. Il semble en effet intéressant de confier au Conseil d'État le soin d'établir une liste d'informations non compromettantes pour la sécurité nationale, mais dont la divulgation entre dans le cadre du droit à l'information. Cela paraît nécessaire au regard de certains scandales touchant des entreprises françaises ayant des intérêts en France et à l'étranger. Pour n'en citer qu'un, on peut s'interroger sur le cas de Lafarge, dont il a été question dans nos débats hier soir. Soupçonnée de financements plus ou moins directs à des organisations terroristes, cette entreprise est-elle prestataire pour l'État en matière de défense nationale ? Cette question nous semble légitime.

Néanmoins, je rappelle que l'article 26 vise justement à mettre en place un dispositif exceptionnel pour les marchés de défense et de sécurité, parce que nombre d'entre eux présentent une sensibilité particulière,

de revient des marchés publics. Il s'agit d'obtenir des titulaires de marchés publics, si besoin par des contrôles sur place, l'ensemble des renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet d'un marché.

qui contribuent significativement aux dépenses d'exécution du marché public et non plus seulement le titulaire du marché. Elles pourront donc inclure les sous-contractants, les filiales et les maisons mères. Deuxièmement, ces enquêtes de coûts pourront porter sur des marchés publics qui n'ont pas été conclus sans mise en concurrence lorsque ces marchés ont pour objet des prestations complexes et d'une durée supérieure à cinq ans. ces enquêtes de coûts pourront être réalisées avant même la notification d'un marché conclu sans mise en concurrence, afin de permettre aux services du ministère d'apprécier le plus en amont possible la pertinence des prix proposés et de négocier ainsi de façon plus efficace. L'élargissement de ce dispositif d'enquêtes de coûts doit permettre de mieux s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics et d'apprécier de façon plus objective l'efficacité des dépenses

le dispositif que vous proposez est assez intrusif pour les entreprises concernées et peut poser un certain nombre de difficultés pour ce qui est du secret des affaires et même de la liberté d'entreprendre.

pour explication de vote. Dans un budget programmé important comme celui-ci, la maîtrise des dépenses reste indispensable. La capacité de mener des enquêtes et des analyses de coûts est une mesure qui nous oblige, oblige, nous, parlementaires, et vous, madame la ministre, quand il est question d'argent public. La Cour des comptes, dans son rapport de février 2013, estimait que des économies importantes pouvaient être obtenues en exerçant une pression plus importante sur les fournisseurs ceux-ci sont relativement peu nombreux, voire en situation de monopole ou de quasi-monopole, et lorsque les marchés sont fréquemment passés selon des procédures négociées sans mise en concurrence et pour des durées longues. Le code des marchés publics autorise déjà ces enquêtes sur les coûts de revient, mais la Cour des comptes avait constaté un manque de moyens humains pour les engager et des négociations trop tardives. Elle avait recommandé notamment de renforcer et de renforcer et de professionnaliser les effectifs d'acheteurs des structures des armées chargées de la maintenance. Le mouvement a été engagé sous le quinquennat précédent puisque, dans son rapport de 2017, la Cour des comptes a constaté que la capacité de négociation de l'État auprès des industriels s'était améliorée

En résumé, nous avons avancé, et nous sommes tout à fait favorables à un renforcement de la capacité du ministère des armées à mieux maîtriser les coûts de ses achats, que ce soit pour la maintenance ou l'achat des équipements. Nous voyons dans votre amendement, madame la ministre, une étape supplémentaire. Je mets aux voix

qui représente tout de même un tiers du parc immobilier de l'État. Alors que les besoins sont en hausse constante, le constat est inquiétant. Il l'est d'autant plus que, malgré cette loi de programmation militaire et la montée en charge des dépenses de défense, il n'est pas sûr que les 2,5 milliards d'euros diagnostiqués par notre collègue Dominique de Legge seront disponibles, et suffisants, d'ici à 2023. Pourtant, l'État maintient sa stratégie de vente du parc immobilier en vue de réduire les dépenses publiques. Il a même conscience que des infrastructures laissées à l'abandon ont été remplies en urgence, notamment depuis la réactivation de l'opération Sentinelle, et sont aujourd'hui en vente à prix réduit si les nouveaux propriétaires s'occupent des travaux de mise en conformité. L'État ne semble pourtant pas en tirer les conclusions nécessaires. l'avancée d'un projet de service national universel dont les contours restent flous fait craindre une nouvelle dégradation des conditions d'hébergement et de vie des soldats. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ! On ne parle pas ici d'infrastructures exceptionnellement occupées, mais de lieux de vie quotidiens. Il est vrai qu'on ne peut pas partir du principe que chaque bâtiment vendu aurait pu servir de lieu d'hébergement, mais je pense sincèrement qu'il faut se poser la question de la réaffectation de ces infrastructures dans un grand plan de réinvestissement pluriannuel du parc immobilier de défense.

favoriser les recettes et les ressources nouvelles pour nos forces armées tant les besoins sont grands. l'article 27 proroge jusqu'en 2025 le régime dérogatoire au régime habituel de cession des biens immobiliers

vente. Nous avons la volonté de faciliter l'action du ministère lorsqu'il veut vendre ses biens, non pas pour un coût inférieur- d'autres amendements nous permettront de revenir sur ce point -, mais pour

des armées est propriétaire d'un grand parc immobilier, qu'il gère de façon active, ce qui donne lieu à un certain nombre de cessions. Ces cessions peuvent bénéficier à des collectivités territoriales pour lesquelles la récupération de ces terrains contribue à la bonne utilisation du foncier public. Le patrimoine immobilier du ministère se voit soumis un mécanisme que vous connaissez bien, du nom de la ministre qui l'a institué, la « décote Duflot », visant à favoriser la mobilisation du foncier public pour accroître l'offre de logements et participer à l'objectif général de cohésion des territoires et de la politique du logement. L'article 28 remet en cause, à la faveur de la loi de programmation militaire, un dispositif général qui s'applique au ministère des armées, mais également bien au-delà du périmètre de ce ministère. J'en

celui où le ministère des armées pourrait récupérer, sous forme de mise à disposition, 100 % des logements qui passeraient par le canal de ce mécanisme. On peut évidemment discuter de la politique immobilière de l'État dans le cadre de la loi de programmation militaire, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait sa place.

que ce soit le lieu pour procéder à des ajustements tout à fait significatifs dans le cadre d'une politique du logement plus globale. Pour cette raison, je vous demanderai de bien vouloir adopter cet amendement de suppression. Quel est l'avis de la commission ? Nos collègues ont

la réalisation de logements sociaux et permettant d'appliquer une décote allant jusqu'à 100 % de la valeur vénale du prix des terrains ou des biens immobiliers cédés par l'État, moyennant une réservation gratuite de 10 % de ces logements au profit des logements sociaux. Lors de la révision de la loi de programmation militaire de 2015, le Sénat, sur l'initiative de notre commission, avait déjà limité le taux de la décote à 30 % pour les terrains occupés par le ministère de la défense, mais cette disposition a été abrogée.

pour les finances du ministère des armées. Scandaleux ! Tout cela serait excessivement positif si, en contrepartie, les fameux logements sociaux bénéficiaient à nos militaires. Ils sont mal logés

Madame la ministre, la solidarité gouvernementale est un fardeau lourd. Nous comprenons tout à fait l'esprit de votre amendement,

dure. Les Français connaissent des attentats. Les troupes françaises remplissent un rôle remarquable à travers la mission Sentinelle pour protéger les Français. Vous êtes ministre des armées, vous devez protéger vos hommes et vos femmes. Comme l'a rappelé le président de la commission, il y a un vrai problème de logement de ces troupes. C'est la première raison pour laquelle il est important d'adopter la position de la commission et, bien sûr, de rejeter votre amendement. Il y en a une seconde, évoquée par l'un de mes collègues. En tant que rapporteur du budget des affaires étrangères, je défends la position que rappelait M. Yung, mais avec un état d'esprit contraire. Pour ma part, j'aurais préféré que tout le patrimoine des armées reste aux armées.

juste un élément d'explication pour répondre à notre collègue Richard Yung. Le dispositif que nous avons mis en place vise effectivement à frapper un grand coup, si je puis m'exprimer ainsi. La crise du logement à Paris est en effet très importante, je l'ai évoqué.

une volonté commune d'offrir à nos soldats les logements décents dont ils ont absolument besoin. On peut parler de la situation à Paris, je pourrais parler du Val-de-Marne et des casernes de gendarmerie, chacun pourrait ici évoquer les problématiques qui sont les siennes.

Or l'immobilier constitue une part importante de ces recettes non aléatoires, qui doivent être des recettes réelles. À partir du moment où s'applique la décote Duflot, ce n'est même plus de recettes aléatoires qu'il s'agit puisqu'il n'y a plus du tout de recettes.

se doit d'être sincère et qu'une recette affectée à un budget n'a pas vocation à financer une autre politique. Je ne reprendrai pas tous les autres arguments- ils ont été excellemment développés par les uns et les autres, notamment par le président Cambon -sur la nécessité de loger dignement nos militaires, notamment à Paris.

pour un dispositif qui favorise la réalisation et la mise à disposition de logements sociaux. C'est ce qui a motivé la rédaction de cet article. Je comprends bien que la commission des finances veuille préserver au maximum les recettes

sauf avis contraire, on ne peut pas avoir les deux, c'est-à-dire favoriser les recettes pour le ministère des armées tout en ayant un vigoureux plan de financement du logement social pour les militaires. Pour le coup, si pareille disposition était votée, elle tomberait, me semble-t-il, je le dis modestement devant un éminent membre de la commission des finances, sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Par conséquent, je propose à Dominique de Legge de nous rejoindre et de retirer son amendement, mais surtout de poursuivre ensemble ce combat,

Jusqu'à maintenant, tous les signes que nous attendions, vous les avez refusés. Je pense au débat d'hier sur les OPEX assez curieux de soutenir que du matériel détruit en OPEX, dans le cadre d'une loi que vous-même qualifiez de « loi de réparation », n'a pas vocation à être remplacé. Vous avez refusé l'indexation.

proposée par la commission des affaires étrangères et que je soutiens, vous pourriez faire un geste ? J'attends votre réponse ; en fonction de ce que vous nous direz, je verrai si je retire mon amendement.

ne devrait pas passer par le canal des cessions. Au fond, s'il s'agit d'affecter 100 % d'un bâtiment appartenant au ministère des armées au logement de militaires, pourquoi faudrait-il le céder ?

vous l'avez également rappelé, c'est celui de l'îlot Saint-Germain. Vous avez eu la délicatesse d'indiquer que nous avions trouvé, à notre arrivée, un certain nombre de décisions déjà prises sur ce dossier.

je l'ai indiqué à plusieurs reprises devant la Haute Assemblée, la politique du logement est l'une de nos priorités et nous l'avons déjà partiellement prise en compte dans le cadre du plan Famille, que j'ai eu l'honneur de présenter devant vous. vous. Monsieur de Legge, puisque vous êtes le représentant de la commission des finances et que vous me chatouillez, si je puis dire, sur la question de la sincérité de ce projet de loi de programmation, je répéterai simplement ce que j'ai dit hier à la tribune et que vous n'avez, me semble-t-il, que partiellement repris : les recettes exceptionnelles qui pourraient résulter de cessions, avait été prévu dans les précédentes lois de programmation, seront des recettes qui viendront par surcroît et dont l'absence ne remettrait pas en cause

la politique du logement de l'État et ne peuvent pas exclusivement se traiter dans le cadre d'une loi de programmation militaire. Cela étant, je suis très sensible au fait que les sénateurs aient prêté une si grande attention

le législateur avait prévu que, pour bénéficier d'une pension, les victimes civiles de la guerre d'Algérie ou leurs ayants droit devaient avoir la nationalité française. Par cette décision QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a censuré cette condition en la déclarant contraire au principe d'égalité. Le Gouvernement entend donc tirer toutes les conséquences de cette censure, tout en recherchant le juste point d'équilibre entre exigences constitutionnelles, soutenabilité du dispositif et nécessité de regarder résolument vers l'avenir, pour donner un nouvel élan à la relation franco-algérienne. Tout d'abord, le respect des exigences constitutionnelles impose la suppression de la condition de nationalité française, jusqu'alors nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une pension en tant que victime civile de la guerre d'Algérie. Dont acte ! Ensuite, l'équilibre du dispositif suppose que les mêmes dommages ne soient pas indemnisés plusieurs fois. Le présent amendement vise à rendre impossible le cumul de la pension concernée avec toute autre indemnisation à raison des mêmes dommages. Enfin, la nécessité de tourner la page de la guerre d'Algérie et de regarder résolument vers l'avenir suppose de borner le dispositif dans le temps. le temps. Les faits étant désormais anciens, il s'avère en effet difficile d'instruire aujourd'hui les dossiers. Le présent amendement a ainsi pour objet de prévoir qu'il ne sera plus possible de présenter de demandes tendant au bénéfice de la pension à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cette disposition garantit pleinement les droits acquis, notamment pour l'ensemble des étrangers ayant déposé une demande de pension depuis la décision du Conseil constitutionnel. pourront bien sûr prétendre au bénéfice de la pension, sous réserve de démontrer que les dommages physiques subis sont imputables à la guerre d'Algérie et qu'eux-mêmes n'ont pas participé, directement ou indirectement, à l'organisation ou à la perpétration de ces violences. Le Gouvernement entend ainsi donner son plein effet à la décision du Conseil constitutionnel et affranchir la relation franco-algérienne des épisodes douloureux du passé. Quel est l'avis de la commission

Cela a été rappelé, plus de cinquante ans après la guerre d'Algérie, il existe aujourd'hui deux catégories de supplétifs : ceux de statut civil de droit local et ceux de statut civil de droit commun. Ces derniers sont actuellement privés de l'allocation de reconnaissance, d'un montant de 3 663 euros. Or 74 d'entre eux, parfaitement identifiés, avaient déposé leur demande entre février 2011 et décembre 2013, période durant laquelle ils étaient éligibles en raison d'une censure constitutionnelle consécutive à une précédente décision QPC. La quasi-totalité d'entre eux, bien souvent âgés et dans des situations précaires, ont été déboutés, voire découragés d'engager des recours contentieux contre les refus de l'administration. Ceux qui l'ont fait ont d'ailleurs eu gain de cause. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Bruno Gilles afin de réparer cette injustice, mais l'Assemblée nationale était revenue dessus.

selon qu'ils étaient arabo-berbères ou de souche européenne, le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 4 février 2011, a considéré que la condition de nationalité était contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens en 2013, en annulant les dispositions qui réservaient le bénéfice de l'allocation de reconnaissance

ouvrant ainsi la voie à l'indemnisation de ceux qui ont déposé une demande d'allocation entre le début de l'année 2011 et la fin de 2013. Mais l'administration est restée sourde à ces demandes. Notre amendement vise donc à permettre aux membres supplétifs

Les explications qui ont été données à la fois par nos collègues Pascal Allizard, au nom de Jean-Pierre Grand, et Jean-Claude Requier ont bien éclairé la Haute Assemblée. Nous avons à prendre une décision dont la dimension humaine

pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a en revanche exclu les membres de formations supplétives de droit commun, c'est-à-dire les personnes d'origine européenne. Le législateur a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d'intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser. évoquent le cas particulier des personnes ayant formé une demande d'allocation de reconnaissance avant le 19 décembre 2013, date d'entrée en vigueur de la LPM 2014-2019, qui a introduit cette distinction selon le statut civil des supplétifs. Dans sa décision QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a réglé le cas de ces personnes, en jugeant que le critère de statut civil ne pouvait justifier le refus d'une demande présentée avant le 19 décembre 2013. Cette décision se suffit donc à elle-même et n'appelle aucune modification de la loi. Les demandes de ces supplétifs de droit commun

une fois de plus, l'égalité de traitement et de reconnaissance de la République envers ceux qui se sont battus pour elle. Nous vous proposons,

La Nation a un devoir de justice envers les membres des forces supplétives en Algérie, qu'ils soient de statut civil de droit local ou de statut civil de droit commun. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam,

supplétifs. Ils ne sont plus que 74. Alors, qu'attendons-nous ? Qu'ils soient tous morts ? Ce serait vraiment une tache sur l'honneur de notre pays, et je compte vraiment sur mes collègues pour se battre

sera-t-il enfin fait droit aux doléances tout à fait légitimes des représentants des associations patriotiques et de mémoire ?

je le redis, nous ne souhaitons pas inscrire ce principe dans la loi. Je comprends très bien que la succession de mesures législatives et de corrections constitutionnelles ait pu égarer les demandeurs,

Les élus des territoires que nous sommes connaissent bien l'importance de l'engagement des associations combattantes non seulement pour faire vivre le devoir de mémoire, mais aussi pour transmettre les valeurs citoyennes reflétées par notre histoire nationale et par les destinées individuelles. individuelles. Malheureusement, nous savons aussi que le temps ne suspend pas son vol. Les combattants de la guerre de 14-18 sont tous décédés, ceux de la guerre de 39-45 vieillissent, tout comme les anciens d'Afrique du Nord, d'Indochine et d'Algérie.

restrictives. Même si je sais que la création de cette décoration ne relève pas à proprement parler de la loi, je tenais, avec mes collègues cosignataires de cet amendement, à demander de nouveau la création d'une médaille d'honneur du monde combattant.

en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation de l'Assemblée nationale du Québec, conduite par son président, M. Jacques Chagnon. La délégation est accompagnée par notre collègue Jean-Claude Carle, président du groupe d'amitié France-Québec. Elle est en visite d'étude sur le thème de l'intelligence artificielle. Cette visite illustre la dimension économique de la francophonie. La délégation s'est rendue ce matin à Saclay, aux laboratoires LIST du Commissariat à À l'occasion de la récente visite à Paris du Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, ce laboratoire et l'Institut québécois de valorisation des données ont signé, le 7 mars 2018, un protocole d'accord pour le renforcement des partenariats scientifiques et d'innovation entre la France et le Québec. La délégation s'est rendue au Petit-Luxembourg, où elle a été reçue pour un entretien par le président du Sénat, M. Gérard Larcher. Elle se rendra ensuite en Haute-Savoie, visitera deux entreprises, Sigma Composite, filiale du groupe Poma, fabricant français de télécabines, et l'« usine du futur » du groupe Baud Industries, spécialisé dans l'usinage de précision. Puis elle aura des entretiens sur le volet agricole de l'AECG, ou CETA, le développement de la montagne et la politique de l'air et de l'eau. La délégation se déplacera enfin au plateau des Glières et déposera une gerbe en mémoire de l'action de la Résistance. Nous souhaitons à nos homologues québécois de fructueux travaux et la plus cordiale bienvenue au Sénat français

L'actualité des dernières semaines ne fait que confirmer nos craintes. Même si le Président de la République ne s'est pas montré solidaire de Donald Trump à propos de l'accord sur le nucléaire iranien,

l'avis de la commission ?

on observe un déséquilibre entre le nombre de ces tribunaux spécialisés et la quantité de dossiers à traiter.

à ces tribunaux spécialisés pour traiter une requête. C'est là une durée excessive, qui a valu à la France d'être condamnée à plusieurs reprises par le Conseil d'État et par la Cour européenne des droits de l'homme. En outre, on constate un manque de jurisprudence disponible, dû à l'absence d'un système de diffusion dématérialisée. En d'autres

leur reconnaissance. Cependant, il faut être bien conscient de la situation actuelle. Le constat est partagé par tous, et d'abord par les associations : les juridictions spéciales ne sont plus adaptées et leurs délais de jugement sont trop longs, cela parce qu'il est difficile de les réunir, humainement et matériellement.

Pour ma part, je pense qu'il est important d'améliorer une situation qui ne peut plus perdurer : les anciens combattants n'ont plus le temps d'attendre. Certes, les tribunaux administratifs sont encombrés, mais les délais de traitement seront quoi qu'il en soit plus courts

Ce transfert permettra de réduire les délais de jugement et de faciliter l'accès à la jurisprudence, tout en conservant un maillage territorial dense. Je remercie M. Yung d'avoir bien développé Les tribunaux administratifs ont largement fait la preuve de leur indépendance et ils sont parfaitement compétents pour traiter ce contentieux dans le plus grand respect des droits des pensionnés. Cette réforme permettra de garantir un service public de la justice à la hauteur de ce que nous devons aux personnes qui agissent

des dispositions très précises quant au caractère public des audiences et à la représentation des parties à l'audience. En outre, depuis la fin de l'année 2016,

l'introduction de dispositions procédurales spécifiques dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre serait redondante et de nature à engendrer des difficultés d'application inutiles.

L'article 32 pose comme principe que les recours à l'encontre des décisions individuelles prises en application du livre Iet du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont précédés d'un recours administratif, afin de favoriser le règlement amiable des litiges. représentants des pensionnés au sein même de la commission chargée de l'examen du recours est un élément important de la réforme des contentieux des pensions militaires d'invalidité. Mais il est nécessaire d'éviter que cette commission

pour ouvrir la possibilité de déterminer par décret en Conseil d'État des exceptions au principe du recours administratif préalable obligatoire pour certaines décisions, en fonction bien sûr de l'objet du litige. Les exceptions seront, par définition, résiduelles. Ainsi, à ce stade, le Gouvernement n'envisage d'exclure du champ du RAPO que les litiges relatifs aux pensions des victimes civiles de la guerre d'Algérie, visées à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour lesquels la présence de représentants d'associations d'anciens combattants paraît moins nécessaire.

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme vous le savez, la réforme du contentieux des pensions militaires d'invalidité inquiète fortement les associations d'anciens combattants. Nous sommes nombreux à avoir été interpellés

Les anciens combattants sont attachés à l'existence de ces tribunaux, qui est liée à la spécificité du droit à réparation. Leurs décisions ont engendré une jurisprudence adaptée. Celle-ci est garantie par leur composition un magistrat professionnel de l'ordre judiciaire, un assesseur médecin expert, souvent au fait de la traumatologie de guerre, et un pensionné au titre des pensions militaires d'invalidité. Ce transfert est sans doute sous-tendu par la volonté de rationaliser la carte judiciaire, ce que l'on peut comprendre, mais comment être sûr que les dossiers des anciens combattants seront mieux traités, et plus rapidement, devant les tribunaux administratifs, qui ont des compétences générales et qui ont beaucoup à faire par ailleurs ? En outre, le manque d'oralité dans la procédure administrative ne risque-t-il pas

le caractère largement oral de la procédure, la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, la mise en oeuvre d'une mission de conciliation ou encore la tenue de l'audience à huis clos à la requête du demandeur. Mon groupe, très attaché

d'État. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant que le taux d'invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle-ci. L'introduction d'une disposition prévoyant que le taux d'invalidité en matière de pensions militaires d'invalidité devrait être déterminé à la date de la demande de pension ne traduit qu'imparfaitement la jurisprudence du Conseil d'État.

Or la gêne fonctionnelle ne peut pas être jugée entièrement au moment de l'instruction première du dossier. L'application conjointe de ces deux critères peut ainsi conduire le juge administratif à ne pas systématiquement retenir la date de demande de la pension comme date de référence

l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Cette ordonnance renforce la contribution du service de santé des armées

Si un conflit à grande échelle devait se produire, il ne commencerait pas par la mise en oeuvre d'armes traditionnelles, mais par une cyberattaque et par l'espace. Dans son discours sur l'état de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker a déclaré que les cyberattaques sont plus dangereuses pour la stabilité des démocraties que les chars et les fusils. Le cyberespace est aussi devenu le lieu de la confrontation informationnelle. Certains pays nous y livrent une guerre au quotidien. Certaines puissances utilisent les moyens numériques pour mener des actions massives et répétées de désinformation et de propagande. de nouvelles techniques mises au service de vieilles tactiques éprouvées visant à manipuler l'opinion publique et à affaiblir les démocraties. Chacun a pu découvrir, avec l'affaire Cambridge Analytica, de quelle manière une puissance étrangère avait pu influencer l'élection américaine.

Notre commission a souhaité que la manipulation de l'opinion publique par l'utilisation massive des médias numériques et des réseaux sociaux, avec pour objectif l'altération du fonctionnement normal des institutions démocratiques, soit prise en compte dans le rapport annexé à la loi

ce champ de réflexion sans attendre, car notre résilience est régulièrement éprouvée, notre vulnérabilité potentiellement élevée et notre arsenal de protection très faible. Si les réponses ne sont probablement pas toutes militaires, il s'agit néanmoins d'un véritable enjeu de sécurité nationale. N'attendons pas un 11-septembre de la « cyber pour comprendre que les démocraties doivent s'allier sans tarder pour combattre un ennemi qui se joue des frontières et cherche à les détruire de l'intérieur. La parole

l'attention à porter, au-delà du volume, au profil des militaires envoyés à Djibouti. Notre mission a mis en évidence le rôle crucial que jouent les familles de militaires dans la présence française sur place, à travers par exemple la situation du lycée français. Nous avons appris qu'il était plus coûteux, pour votre ministère, d'affecter des militaires en mission longue, surtout s'ils font venir leur famille. Sur le plan interministériel du rayonnement de notre pays, il faut toutefois mesurer que la présence des familles est un outil d'une efficacité considérable, et relativement peu coûteux,

dans le domaine « cyber ». Un certain nombre de grandes démocraties ont expérimenté à leurs dépens la menace que peuvent représenter les cyberattaques en termes de mise en cause des fondements mêmes de la démocratie.

Fonds européen de défense, création de forces d'intervention communes : Paris ne ménage pas ses efforts pour faire émerger une défense fédérale au niveau européen.

une position européenne et une position atlantique dans ce même cadre ? La création d'un nouvel organe de défense pourrait créer une confusion semblable à celle qui existe déjà entre l'ONU et l'OTAN.

Cette inquiétude est d'autant plus prégnante que le Fonds européen de défense est fortement convoité, nous semble-t-il, par les grands groupes états-uniens de défense. Second écueil : le proto-fédéralisme qu'implique une Europe de la défense. Quelle force de gouvernance, alors même que l'Union

Cette situation nous fait craindre une incapacité de la France à maintenir un semblant d'indépendance industrielle et de défense et un nouveau drame humain dans l'emploi industriel.

Aujourd'hui, il nous faut réaffirmer le caractère solidaire de l'Union européenne, sans remettre en cause le principe de souveraineté des peuples et des États,

Israël, qui occupe les territoires palestiniens au mépris du droit international. L'emploi sert très souvent de paravent magique à la volonté de développer l'exportation d'armements. Pourtant, l'emploi industriel dans ce secteur est en baisse constante, malgré la multiplication des contrats, du fait de la libéralité de la France en matière de transferts de compétences et de recours au travail détaché.

Cet amendement vise à mentionner explicitement dans la loi les articles 26 et 51 de la Charte des Nations unies. Aujourd'hui, le choix de la France de faire de l'exportation d'armements une variable d'ajustement de sa balance commerciale tend à rompre l'équilibre entre ces deux articles. De fait, c'est bien un équilibre qu'il faut trouver entre la nécessaire raréfaction des armes en circulation et le droit des États à assurer leur sécurité.

satisfaire leurs besoins en matériels de guerre ou de police. Toutefois, la France ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités dans la prolifération des armements.

pose par ailleurs la question des menaces. On constate aujourd'hui un véritable cercle vicieux, puisque, du fait de conflits, de pressions

travailler à conforter l'Europe de la défense. Nous ne sommes pas des rêveurs : nous savons bien qu'elle est très difficile à constituer. J'ai dit moi-même qu'elle devrait commencer par des achats communs, qui faciliteraient l'interopérabilité entre les forces armées. Il y a un long chemin

tout transfert ou vente d'armes à des pays sous embargo. Nous respectons bien évidemment les procédures de notification

qui consiste, au fond, à éliminer toute référence à la politique européenne. Au contraire, le Gouvernement fait de la coopération européenne et de la construction d'une Europe de la défense,

l'idéologie à laquelle il se réfère. De fait, assimiler exclusivement le terrorisme au terrorisme djihadiste me semble réducteur.

des inquiétudes du côté iranien et quelques espoirs du côté coréen. En effet, le rapport annexé évoque le caractère contraignant de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien. Hélas,

Alors que l'Union européenne se mobilise pour déminer la situation, les États-Unis ont encore accentué leur position hier, par la voix de leur nouveau secrétaire d'État, Mike Pompeo. Celui-ci a fait une nouvelle démonstration de force face à l'Iran, en dressant une liste de douze conditions à respecter, dont certaines sont sans rapport avec le programme nucléaire iranien et beaucoup sont irréalisables. tend également à la prise en compte de la nouvelle donne concernant la Corée du Nord, qui, sans abandonner complètement son programme nucléaire, promet le gel des essais et la destruction des sites. Nous avons choisi une terminologie qui atténue la rédaction actuelle de l'alinéa 25, tout en restant prudents dans le choix des mots, car la vigilance s'impose toujours sur la question de la prolifération nucléaire dans ce pays.

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, je ne veux évidemment pas répondre à la place du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, mais, comme vous l'avez indiqué, la France, avec ses partenaires européens, en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont signataires du traité de Vienne, a rappelé son attachement à poursuite de la mise en oeuvre de ce dernier. La réunion qui s'est tenue à Bruxelles en présence de Mme Mogherini, qui est également partie prenante à cet accord au nom de l'Union européenne, a confirmé l'unité européenne autour de cette volonté de poursuivre l'application du traité de Vienne, malgré les décisions prises par les Américains. Pour l'Iran, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les conséquences économiques du retrait américain. Pour l'Europe,

du traité de Vienne pourrait avoir sur l'ensemble de la région. Cela nous conduirait très loin, puisque l'Iran est très influent au Moyen-Orient. Le président Macron a été amené

appelé l'attention sur le fait que les agissements de l'Iran en matière balistique et son influence au Moyen-Orient devaient faire

: La parole est à M. Joël Guerriau. Les moyens dédiés à la fonction « prospective » du ministère des armées ne sont pas évoqués dans le rapport annexé, alors qu'ils apportent une contribution importante à la fonction stratégique « connaissance et anticipation la stratégie, la DGRIS, en tant que coordinateur du réseau d'universités et de spécialisés dans la défense, devront être renforcés. La société civile participe en effet pleinement à la fonction « connaissance et anticipation » des armées, par l'intermédiaire d'une recherche stratégique et prospective à la fois dynamique et innovante.

missions. Les gouvernements successifs se sont lancés dans une politique de réduction des dépenses publiques. Avant, on déterminait les besoins, puis on établissait le cadre ; aujourd'hui, on fixe le cadre, et tout ce qui en dépasse est privatisé ou abandonné.

du Gouvernement ?

effrayante. L'arsenalisation de l'espace constitue aujourd'hui un véritable enjeu et un nouveau risque que la France doit appréhender. C'est pourquoi nous souhaiterions inscrire dans la loi que notre pays invitera sous peu ses partenaires à la table des négociations, dans le cadre de l'ONU,

Il nous semble essentiel que la France inscrive noir sur blanc son engagement à ne pas intervenir à l'étranger sans mandat de l'ONU.

elle ne peut pas lier sa capacité d'intervention aux décisions d'une organisation internationale, quelle que fût la qualité de celle-ci. J'observe au passage que, tous gouvernements confondus, notre pays fait en sorte d'assumer ses responsabilités au sein du Conseil de sécurité et d'intervenir la plupart du temps sous mandat de l'ONU.

d'autant que l'accolement des missions de contre-terrorisme et de contre-insurrection tend à assimiler terrorisme et insurrection. Or il ne s'agit pas de la même chose.

La contre-insurrection devrait plutôt relever des missions de police. De fait, dans le cas hypothétique où des militaires français seraient engagés contre des insurgés français, on passerait d'une insurrection à une véritable guerre civile.

... Même si la France peut théoriquement intervenir à la demande du pays concerné, la prudence voudrait qu'elle s'abstienne. Il me semble donc essentiel d'éviter que le recours à l'armée soit la réponse apportée à une insurrection,

et sécurisant, pour les armées, d'attendre l'issue des élections présidentielles et législatives de 2022 pour procéder à l'actualisation de la loi de programmation militaire.

Pour rappel, un rapport de l'Assemblée nationale en date du 16 décembre 2015 soulignait déjà le niveau critique des stocks au regard du rythme des frappes réalisées par nos armées. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée ; elle s'est même aggravée, avec l'intensification des opérations au Levant. dans ce rapport, à l'époque, le temps des industriels ressortissant au temps long, il a fallu faire appel aux munitions de nos alliés. Depuis, il semble que la problématique ait peu évolué, alors que ce sujet d'importance stratégique pour les forces a été mis en lumière par la Revue stratégique Il me semblerait donc logique que la LPM prenne en considération cette problématique, afin que le ministère des armées apporte des solutions concrètes, visant à assurer la disponibilité constante des munitions et l'accroissement de leur volume.

En témoigne la disparition de la filière « bombe » en France, qui impose à notre pays l'achat de corps de bombe, sur étagère et sur liste d'attente, auprès d'autres États. Comme pour les munitions de petit calibre, la France devrait réfléchir à la reconstruction d'une filière nationale pour combler cette lacune.

et à s'assurer de la disponibilité de filières d'approvisionnement fiables et efficaces. La question de l'autonomie que vous soulevez, madame la sénatrice, n'a pas forcément de sens pour tous les types de munitions.

mais les prévisions ont été mises à mal par la volonté politique de réduction des dépenses publiques, et donc des effectifs de fonctionnaires. De fait, aujourd'hui, le développement de la réserve vise plus à en faire une force palliative qu'une force de soutien. À ce titre, il faut citer le cas assez symptomatique du service de santé des armées, qui mobilise déjà près de 3 000 réservistes, représentant 10 % du contrat opérationnel. Je ne suis pas persuadée que le recrutement prévu dans la loi de programmation militaire soit suffisant pour, à la fois, couvrir les besoins en femmes et hommes engagés et refaire de la réserve une force de complément exceptionnelle,

d'être affectés temporairement à un emploi administratif. Cet aménagement leur permettrait de s'occuper au mieux de leur enfant sans renoncer à leur carrière ni à leurs revenus et de bénéficier d'horaires de travail fixes et réguliers. Actuellement, les militaires peuvent demander un congé de présence parentale. Celui-ci est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins pénibles. Dans de nombreux cas, les horaires de travail atypiques des militaires sont difficilement conciliables avec leur vie familiale. Ce constat est d'autant plus vrai pour les familles dont les deux parents sont des militaires et pour les militaires déployés à l'étranger, en opération extérieure. cette mesure permettrait aux militaires concernés de conserver leur emploi, tout en bénéficiant d'horaires stables, plus compatibles avec les besoins de leurs enfants. Elle serait susceptible d'améliorer les conditions de vie de nombreux militaires pères ou

annexé, qui est ainsi rédigé : « En particulier, à Paris, la cession d'une partie du site du Val-de-Grâce sera reconsidérée au regard de la nécessité, pour le ministère des armées, de conserver une emprise d'envergure à l'intérieur de Paris. » Nous avons déjà longuement évoqué cette question. La cession du site du Val-de-Grâce a été décidée, actée dans son principe, même si elle n'est pas encore effective. Je rappelle que des recettes sont attendues au titre de cette cession. Même si

à être cédé et que les recettes afférentes devront être affectées au ministère des armées. Pour cette raison, je demande la suppression de cet alinéa du rapport annexé.

ne se substitueront pas aux crédits d'infrastructures programmés, mais viendront consolider une réalisation de la programmation équilibrée et conforme aux ambitions fixées par la LPM. » J'avoue avoir un peu de mal à comprendre que ce qui était faux voilà une heure soit maintenant devenu vrai ... Vous avez même ajouté tout à l'heure

Le rapport d'information de Mme Geneviève Gosselin-Fleury soulevait déjà la complexité, sur les plans structurel, fonctionnel et financier, de la garde des enfants pour les militaires. Les parents, en particulier lorsque les deux conjoints sont militaires, ont de grandes difficultés à trouver un mode de garde adapté aux exigences de leur profession. Ce souci quotidien est encore accru pour les familles monoparentales ou pendant l'absence du conjoint ou de la conjointe, qui peut durer des mois, voire une année. Les horaires atypiques et les absences liées aux missions des parents militaires engendrent des difficultés pour la garde des enfants. Si le ministère a mis en place le plan « petite enfance 2015-2019 », en finançant des établissements et en prenant en charge une partie de l'accueil, il n'existe pas de solution unique en fonction de la localité, de l'éloignement du lieu de résidence, des horaires de travail, de la composition de la famille, de sa capacité financière ou du mode de transport. Il est donc indispensable que les militaires puissent avoir

L'allégement des démarches doit aussi être envisagé. En effet, les familles sont trop souvent découragées par le volume des formalités administratives. Le présent amendement vise à généraliser les offres de garde adaptées aux contraintes particulières liées à l'exercice professionnel des militaires. C'est aussi un moyen de fidéliser

qui en souffrent. Pourtant les conséquences, on le sait, peuvent être graves pour le militaire, sa carrière, ses frères d'armes et sa famille. Ces blessures peuvent briser des vies. Aussi est-il impératif de renforcer le dépistage au sein même des régiments et, ensuite, de rendre accessible un accompagnement, un suivi spécifique des soldats affectés par ces troubles. Dans l'histoire des opérations extérieures et intérieures françaises, les années 2012 à 2017 auront été particulières, marquées par un niveau de sollicitation extrême et l'usure des personnels. Je crois que la reconnaissance de la Nation passe aussi par le soutien à ses soldats. Je salue bien évidemment le travail mené

La cellule Thémis, indépendante des hiérarchies, travaille en liaison avec les inspecteurs généraux des armées. Elle est tenue à une obligation de discrétion et de confidentialité. Elle observe la plus stricte neutralité. Elle est chargée d'examiner les cas de harcèlement, de discrimination, de violences sexuelles ou à connotation sexiste, ou liées à l'orientation sexuelle des personnes, et de veiller à ce que les infractions avérées soient sanctionnées à hauteur du préjudice infligé. La cellule peut être saisie de diverses façons. Chaque personnel du ministère des armées, qu'il soit civil ou militaire, femme ou homme, victime ou témoin d'une infraction, peut la saisir.

La cellule Thémis offre une écoute adaptée et attentive aux victimes, par des interlocuteurs et interlocutrices dédiés et formés en conséquence. Un accompagnement pluridisciplinaire, juridique, social et professionnel est mis à disposition des victimes. Un suivi des enquêtes disciplinaires et une vérification de la proportionnalité des sanctions sont également assurés. Le ministère est invité à poursuivre et à accroître son action en interne de sensibilisation, d'information et de formation dans le cadre de sa lutte contre les violences sexuelles et sexistes,

Alors je n'ai rien dit

: La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement vise à introduire, dans la partie du rapport annexé consacrée à la gestion des ressources humaines, un titre permettant de faire apparaître de manière lisible un certain nombre de développements concernant la politique du ministère des armées en matière de lutte contre les discriminations. Les discriminations de toute nature, notamment les discriminations sexuelles, sont une réalité qu'il ne faut pas occulter ni négliger. De nombreux efforts sont réalisés dans ce sens, notamment la création de la cellule Thémis, qui permet à chaque personnel du ministère des armées, civil ou militaire, victime ou témoin de harcèlements, de discriminations ou de violences sexuelles au sein du ministère de signaler ces faits. En introduisant un alinéa dédié à la lutte contre toutes les formes de discriminations, nous encouragerions le ministère à poursuivre ses efforts dans ce domaine.